Monsieur le président,

les crédits de paiement alloués à cette mission s'élèvent à 27 milliards d'euros. Ils progressent de plus de 500 millions d'euros. Ces augmentations doivent être mises en regard des annulations de crédits prévues dans le projet de loi de finances rectificative pour 2018, qui se montent à plus de 200 millions d'euros sur cette mission. Ce que la loi de finances donne, la loi de finances rectificative peut le reprendre en gestion, ce qui limite la portée de notre vote de ce jour ! Exactement ! Le budget de l'enseignement supérieur s'inscrit, cette année, dans la trajectoire dessinée par la loi de finances 2018. Les programmes 150, « Formations supérieures et recherche universitaire », et 231, « Vie étudiante », connaissent une légère progression de plus de 1 %, soit 173 millions d'euros en crédits de paiement. Ce budget est globalement satisfaisant, madame la ministre, dans le contexte budgétaire actuel. De plus, il faut prendre en considération les crédits consacrés à l'enseignement supérieur et à la recherche dans le Grand plan d'investissement, qui s'élèvent à 645 millions d'euros. Je partage les principales orientations de la politique sous-tendant ce budget, en particulier, le plan Étudiants et l'importance accordée à l'orientation- c'est en orientant mieux les étudiants que l'on réduira l'échec en licence, qui touche 40 % d'entre eux -, ainsi que l'insertion professionnelle des jeunes. Voilà pour le positif. Mais j'ai aussi quelques réserves, madame la ministre. J'observe, cette année encore, que les dépenses salariales contraintes ne sont pas intégralement budgétées, et ce dans une fourchette allant de 50 millions à 100 millions d'euros. Il est insupportable de ne pas prévoir une dépense pourtant certaine. Le glissement vieillesse-technicité, le GVT, des établissements- une dépense obligatoire -ne pourra pas être couvert. Par ailleurs, de nombreux emplois pourtant budgétés ne seront pas créés puisqu'ils servent de variable d'ajustement. Ce n'est pas une bonne méthode, et cela réduit la portée des moyens annoncés. S'agissant des dotations des universités, la subvention pour charges de service public notifiée à chaque établissement est aujourd'hui encore presque intégralement déterminée à partir du montant de la notification de l'année précédente, à laquelle sont appliqués différents ajustements, très marginaux puisqu'ils n'excèdent pas 5 %. Je souhaite, madame la ministre, que votre administration s'oriente vers un pilotage plus fin des dotations aux opérateurs, tenant compte, notamment, de la stratégie et des enjeux propres à chacun d'eux. Les ressources propres de ces universités ne représentent, en moyenne, que 16 % de leurs dépenses de fonctionnement, ce qui est tout à fait insuffisant. On espère que la valorisation de la recherche pourra faire évoluer la situation. Les frais d'inscription demeurent extrêmement faibles. M. le Premier ministre a annoncé que les étudiants non européens pourraient voir leur cotisation augmenter substantiellement, potentiellement de 170 euros à 2 700 euros, récent rapport, la Cour des comptes recommande d'augmenter également les frais d'inscription pour les étudiants français, du moins en master et en doctorat, mais à des niveaux moindres. après année, je milite pour que l'on améliore la situation des étudiants, en augmentant les frais d'inscription. On accepte aujourd'hui plus facilement de payer une cotisation à un club de sport, dont l'effet ne sera pas le même sur l'avenir des jeunes

ces nouvelles ressources seront, et devront l'être, de la responsabilité des universités, pour leur montant comme pour leur affectation. Madame la ministre, entendez-vous néanmoins faire des préconisations pour que ces sommes soient mises au service des étudiants, de leur environnement, de la pédagogie ? Il ne serait pas normal qu'elles servent à pallier l'absence de financement par l'État pour, par exemple, le GVT. Je souhaite, sur ce point, avoir des assurances Le soutien à l'enseignement supérieur privé demeure trop limité, de mon point de vue. Le montant moyen de la subvention de l'État par étudiant a diminué de 45 % entre 2008 et 2018. et 2018. C'est d'autant plus préjudiciable que les établissements d'enseignement supérieur accueillent un nombre croissant d'étudiants. Un étudiant inscrit dans un établissement d'enseignement supérieur privé d'intérêt général, un EESPIG, est aujourd'hui soutenu par l'État à hauteur de 600 euros, en moyenne, alors que le coût par étudiant dans le secteur public s'élève à plus de 9 000 euros, et l'économie que représentent ces 100 000 étudiants pour le budget de l'État s'élève donc à environ 800 millions d'euros. mes chers collègues, la commission vous propose d'adopter un amendement tendant à augmenter la dotation allouée à ces établissements, dont certains éprouvent de réelles difficultés, et ce d'autant plus si certaines municipalités se désengagent. Les Les crédits du programme 231, « Vie étudiante », connaissent des changements modestes pour 2019. Le projet de loi de finances introduit la contribution vie étudiante et de campus, la CVEC, dans la liste des taxes affectées, plafonnant son produit à 95 millions d'euros. Dans la mesure où la collecte de 2018 semble d'ores et déjà s'établir autour de 115 à 120 millions d'euros, une vingtaine ou une trentaine de millions d'euros collectés sur le revenu des étudiants pourraient ainsi abonder le budget de l'État et participer à l'équilibre des finances publiques. J'estime, madame la ministre, que l'argent ainsi collecté doit être intégralement affecté à la vie étudiante et que le plafond de cette taxe affectée doit être réévalué et amendé dès le projet de loi de finances pour 2019.

tous les étudiants paieront cette contribution, y compris ceux qui sont inscrits dans des EESPIG, ces derniers recevront seulement 20 euros en retour, contre 40 euros pour les étudiants des établissements publics. Je ne comprends pas cette inégalité de traitement, madame la ministre, et j'aimerais que vous nous disiez ce que vous comptez faire pour y remédier.

en 2019, soit une hausse de 330 millions d'euros- 2,9 % -par rapport au budget 2018. Le budget pour 2019 s'inscrit ainsi dans la trajectoire dessinée pour 2018, avec une forte progression des crédits alloués à ces programmes sur deux ans : de l'ordre de 817 millions d'euros en autorisations d'engagement de 440 millions d'euros en crédits de paiement. Le montant total des crédits alloués aux programmes dépendant du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, c'est-à-dire les programmes 172, « Recherches scientifiques et technologies pluridisciplinaires et 193, « Recherche spatiale », s'établira à 8,8 milliards d'euros, soit une forte hausse de 376,4 millions d'euros par rapport à 2018. Ces programmes captant l'intégralité de la hausse des crédits de la mission, je souhaiterais m'arrêter sur quelques points saillants qui m'ont interpellé au cours des auditions. Tout d'abord, le budget alloué à la recherche spatiale, en progression de 205 millions d'euros, absorbe les deux tiers de l'augmentation des crédits du volet « recherche », pour atteindre 1,8 milliard d'euros. Cette hausse serait destinée à financer les engagements de la France sur le programme Ariane 6, tout en poursuivant l'apurement de la dette française auprès de l'Agence spatiale européenne, l'ESA. Je note à ce sujet, madame la ministre, que la contribution française à l'ESA franchit cette année le cap symbolique du milliard d'euros, en passant de 963 millions d'euros à 1,17 milliard d'euros en 2019. en 2019. Par ailleurs, le relèvement des moyens financiers de l'Agence nationale de la recherche, l'ANR, se poursuit. Avec une augmentation de 86,3 millions d'euros en crédits de paiement, l'agence devrait être en mesure de renouer avec un taux de succès sur les appels à projets supérieur à 15 %. Peut-on pour autant considérer que l'objectif que s'est fixé le Président de la République, à savoir redonner à l'ANR des moyens dignes de ceux de ses homologues étrangers, est atteint ? Assurément pas L'augmentation de son budget doit rester une priorité pour se rapprocher des standards européens en matière de recherche sur projets, avec un taux de succès moyen de 24 %. Cette évolution est d'autant plus nécessaire que nos chercheurs peinent à obtenir des financements européens, comme en attestent les chiffres du programme-cadre Horizon 2020, peu flatteurs pour la France. Enfin, le plan Intelligence artificielle bénéficiera de 17 millions d'euros en 2019, auxquels s'ajoutent 12 millions d'euros en provenance des programmes d'investissements d'avenir, les PIA, pour accompagner la mise en place d'un réseau emblématique d'instituts dédiés à l'intelligence artificielle. Je ne peux que saluer, madame la ministre, les efforts consentis afin de doter la France d'une véritable stratégie en matière d'intelligence artificielle. Je regrette néanmoins que les moyens alloués au plan Intelligence artificielle en 2019 demeurent très en deçà des annonces gouvernementales, d'une part,

S'il faut nous féliciter de toutes ces hausses de crédit, je tiens à rappeler qu'elles se font au détriment des organismes de recherche, lesquels voient leurs dotations diminuer ou stagner. Confrontés à une augmentation considérable de leur masse salariale, ces organismes n'ont souvent d'autre choix que de réduire leurs effectifs, ce d'autant, madame la ministre, que le GVT n'est pas compensé pour eux- Philippe Adnot vient de le préciser. Les directeurs des organismes de recherche m'ont, par ailleurs, signalé plusieurs situations d'impasse budgétaire. Ainsi le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, à un surcoût de plusieurs centaines de millions d'euros dans le cadre de la construction du réacteur Jules Horowitz, tandis que les plans Santé commandés par le Gouvernement à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, l'INSERM, doivent bénéficier des financements adéquats, combinés, d'ailleurs, avec les fonds européens sur certains programmes. À plus long terme, l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer, l'IFREMER, devra faire face à des besoins de financement de l'ordre de 500 millions d'euros pour le renouvellement de la flotte océanographique, sans qu'aucun plan d'investissement à moyen terme ait été élaboré à ce jour. Je note toutefois avec satisfaction que le Premier ministre a annoncé le lancement d'une réflexion à ce sujet, lors du comité interministériel de la mer du 15 novembre. Je ne saurai qu'inviter le Gouvernement à poursuivre dans cette voie, de manière à anticiper au mieux les besoins d'investissement de notre flotte océanographique. Les autres programmes, qui ne dépendent pas du ministère de la recherche et de l'enseignement supérieur, voient leurs crédits stagner ou diminuer en 2019. Ce sera notamment le cas des programmes 192, « Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle 191, « Recherche duale (civile et militaire) », et 186, « Recherche culturelle et culture scientifique ». Deux exceptions à cette tendance morose Le programme 142, « Enseignement supérieur et recherche agricoles », qui porte, notamment, les crédits de l'Institut national de la recherche agronomique, l'INRA, et de l'Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture, l'IRSTEA, voit ses crédits progresser de 2 %. Je voudrais rappeler, à ce sujet, que l'année 2019 sera marquée par la préparation de la fusion de ces deux organismes en un institut unique, qui devrait voir le jour le 1 janvier 2020. Il était temps ! Une enveloppe de 4 millions d'euros supplémentaires est débloquée pour couvrir les besoins engendrés par ce processus. Le programme 190, « Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables » bénéficiera, lui, d'une augmentation de 5,8 millions d'euros. J'attire néanmoins votre attention sur le fait que, en dépit de cette hausse, l'Institut français du pétrole-Énergies nouvelles, l'IFPEN, verra sa subvention diminuer de 4,1 millions d'euros en 2019, puis en 2020. Je voudrais terminer mon intervention par quelques considérations sur le crédit d'impôt recherche, ou CIR. Si cette dépense fiscale représente un coût considérable pour les finances publiques, de l'ordre de 6,2 milliards d'euros en 2019, la plupart des évaluations s'accordent à reconnaître l'existence d'un effet positif. Pour que Pour que la France ne se laisse pas distancer dans la compétition internationale, pour qu'elle reste la cinquième puissance scientifique mondiale, ce soutien à la recherche privée doit être maintenu.

Monsieur le président, madame la ministre, mesdames, messieurs les rapporteurs, mes chers collègues,

budget, il faut absolument réduire les coûts et amplifier l'effort d'innovation dans le domaine des lanceurs. Les États européens doivent également s'accorder sur le principe de « préférence européenne ». Notre souveraineté en dépend. Sur l'Agence nationale de la recherche, l'effort budgétaire mériterait d'être amplifié à l'avenir, pour parvenir à un taux de sélection de 20 % et éviter le découragement des chercheurs. Sur le programme 190, nous appelons à la plus grande vigilance sur la situation de trésorerie de l'IFPEN, qui connaît une baisse continue de sa subvention. Sur le programme 192, la diminution de la dotation servant à financer les aides à l'innovation octroyées par Bpifrance doit cesser. Le plancher de 120 millions d'euros ne devra pas être dépassé. Quant à la suppression du fonds unique interministériel, qui marque un désengagement de l'État dans la politique des pôles de compétitivité, il ne faudrait pas, madame la ministre, qu'elle conduise à l'assèchement financier. Les rôles respectifs de l'État et des régions dans la phase IV des pôles mériteraient aussi d'être clairement définis. J'ai porté une attention particulière à la stratégie nationale pour l'intelligence artificielle. a probablement trop tardé, mais elle a le mérite d'exister. Si le chiffre de 1,5 milliard d'euros sur cinq ans peut impressionner, il est à relativiser, au regard des investissements publics réalisés par les États-Unis et la Chine en rapport à leur poids dans l'économie mondiale. Mais, surtout, 9 % seulement de cette somme sera composée de crédits nouveaux. La mise en oeuvre a déjà débuté en 2018, ce qu'il convient de saluer. Il s'agit dorénavant d'accélérer, car la France ne peut se permettre de perdre plus de temps. Il conviendrait de s'appuyer sur des coopérations bilatérales et de peser sur la définition de la stratégie au niveau européen pour décupler l'impact de la nôtre. Enfin, madame la ministre, il serait bienvenu que, à l'avenir, la ventilation des crédits affectés au plan soit bien précisée dans les documents budgétaires. La parole est à Mme

madame la ministre, mes chers collègues, notre collègue Jean-François Rapin a rappelé les évolutions positives des crédits consacrés à la recherche. Celles-ci ne doivent cependant pas masquer les menaces qui pèsent sur la recherche à moyen terme. Il y a lieu, tout d'abord, de s'inquiéter de la place de plus en plus importante que prennent les financements sur projets dans le budget des opérateurs de recherche. S'ils constituent désormais des ressources complémentaires indispensables, ils ne compensent que partiellement la diminution de la dotation de base dans le temps. Il faut, ensuite, aborder avec lucidité la question du niveau des subventions pour charges de service public ; celles-ci sont à ce jour largement obérées par l'augmentation de la masse salariale, notamment par le coût du glissement vieillesse-technicité. Ces charges salariales élevées, subies et, donc, indépendantes de la stratégie des opérateurs en matière de ressources humaines contraignent un certain nombre d'entre eux à réduire leurs effectifs, dans des proportions parfois importantes. Une telle situation n'est pas tenable à long terme et menace les projets de recherche.

En conclusion, je souhaiterais appeler votre attention sur trois objectifs, qui me semblent prioritaires pour 2019. Le premier objectif est, de mon point de vue, la nécessaire revalorisation salariale des chercheurs et la remise à plat de leur régime indemnitaire. Il y va de l'attractivité du métier de chercheur et de la capacité de la France à tenir son rang dans le domaine stratégique de recherche. Le second objectif est de réussir la fusion entre l'INRA et l'IRSTEA. C'est un beau projet scientifique, qui doit être soutenu financièrement par les deux ministères de tutelle jusqu'au bout. Le troisième objectif est de rétablir un lien de confiance entre l'État et le CEA, et d'éviter que les solutions arrêtées pour limiter le coût des projets de recherche dans le nucléaire ne pénalisent l'ensemble des activités de recherche du Enfin, je ne saurais trop insister sur la nécessité de donner au plateau de Saclay les moyens de ses ambitions. Vitrine française de la recherche et de la formation à l'international, le projet du plateau de Saclay est aujourd'hui menacé dans son développement par l'absence d'infrastructures de transport dignes de ce nom. Il y a urgence à ce que soit construite la ligne 18 du métro du Grand Paris Express. Sous les réserves que je viens d'évoquer, la commission de la culture, de l'éducation et de la communication a émis un avis favorable à l'adoption des crédits de la mission « Recherche et enseignement supérieur ». La parole

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, au sein de la mission interministérielle « Recherche et enseignement supérieur », la MIRES, qui représente tout de même 6 % du budget général de l'État, avec 28 milliards d'euros, le programme 150 est en légère augmentation de 1,2 %. Les 166 millions d'euros de crédits supplémentaires, auxquels il convient d'ajouter un moindre gel des crédits à hauteur de 40 millions sont à mettre en perspective avec l'inflation à 1,7 %, l'augmentation du budget de l'État de 1,9 %- je ne suis pas sûr que ce soit une bonne référence -et, surtout, l'augmentation des effectifs d'environ 2,5 % sur les deux rentrées de 2018 et 2019.

Il est extrêmement regrettable que de telles charges, qui dépendent de décisions prises par l'État, ne soient pas intégralement compensées. En définitive, sur l'enveloppe globale, bien peu servira à améliorer les conditions d'études supérieures, alors même que c'était l'objectif prioritaire annoncé par le Gouvernement. Concernant les établissements privés, j'ai souhaité, comme mon collègue Philippe Adnot, porter un amendement de réévaluation sur trois ans de la contribution aux EESPIG, à hauteur de 1 000 euros par étudiant. Rappelons que, depuis 2000, on constate une augmentation de 62 % des effectifs dans les établissements privés, à comparer à la hausse globale des effectifs de 18 %. Ce coup de pouce est possible en puisant sur le fonds mobilité, curieusement porté à 30 millions d'euros, alors que les crédits consommés cette année ont été très maigres. De même, le plafonnement de la CVEC à 95 millions d'euros interroge, alors que le montant de la collecte à la rentrée, déduction faite des remboursements aux boursiers, s'élève à environ 120 millions d'euros. Près d'un an après l'adoption du projet de loi relatif à l'orientation et à la réussite des étudiants, il conviendra d'observer l'évolution du taux de réussite en licence en trois ans- moins de 30 % aujourd'hui mais aussi de la part des sortants du supérieur sans diplôme, 17 % à l'heure actuelle. Les objectifs du Gouvernement dans ce domaine sont particulièrement mesurés La création de 31 000 places au printemps, puis cet été, dans les établissements de l'enseignement supérieur est de nature à faire face à l'arrivée de nouveaux étudiants. Mais des places vacantes, de l'ordre de 120 000, à l'issue de la procédure Parcoursup ? De même, l'absence d'accompagnement financier de la réforme annoncée des études de santé, qui va pourtant entrer en vigueur à la rentrée de 2019, est aussi surprenante.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable s'est saisie, comme chaque année, du programme 190 de la mission « Recherche et enseignement supérieur », qui soutient les activités de sept opérateurs dans les domaines du développement durable, de l'énergie, des risques, des transports, de la construction et de l'aménagement du territoire. À l'heure de la transition écologique, ce programme revêt une importance fondamentale en tant qu'appui scientifique aux politiques en faveur du développement durable. Ses crédits sont relativement stables par rapport à l'année dernière, ce dont nous pouvons nous réjouir. Mais cette trajectoire globale cache une évolution inégale des subventions allouées aux différents opérateurs. Comme les années précédentes, le principal bénéficiaire du programme reste de loin le CEA, qui reçoit 1,22 milliard d'euros, soit plus de 75 % des subventions pour charges de service public prévues par le programme. C'est la raison pour laquelle je voudrais insister, madame la ministre, sur la nécessité d'accélérer les investissements dans la recherche liée, en particulier, Le CEA mène en effet d'importants travaux sur cette production décarbonée et sur son utilisation dans les mobilités, domaines dans lesquels la recherche française conserve encore une certaine avance. Mais pour combien de temps encore ? Il est donc plus que jamais indispensable d'accélérer l'expérimentation et l'amélioration de la performance des infrastructures de production, mais aussi de stockage et de transport de l'hydrogène. D'autres pays ont récemment accéléré le déploiement de cette technologie : ainsi, l'Allemagne a mis en service son premier train à hydrogène, en Basse-Saxe. Ma deuxième observation portera sur la subvention attribuée à l'IFP qui diminue de plus de 4 millions d'euros, confirmant une tendance à la baisse observée depuis plusieurs années. En effet, la dotation à l'institut est passée de 169 millions d'euros en 2010 à 128 millions, soit une diminution de près de 25 %. Or l'IFPEN soutient de nombreux projets en matière de nouvelles technologies de l'énergie, en particulier en partenariat avec de petites et moyennes entreprises Madame la ministre, lors de l'examen du projet de loi de finances à l'Assemblée nationale, vous avez évoqué un redéploiement de 1 million d'euros en faveur de l'IFPEN. Pouvez-vous nous confirmer cette décision et nous en préciser les modalités ? Pour conclure, je voudrais insister sur l'impérieuse nécessité de maintenir les fonds alloués au programme 190. Au vu des actions menées par les différents opérateurs, ces ressources contribuent non seulement à la décarbonation de notre économie, mais également à sa compétitivité face à une à sa compétitivité face à une concurrence internationale de plus en plus rude, y compris en matière d'énergies renouvelables et de transition écologique. Il est donc vital de maintenir un engagement financier à la hauteur des enjeux. Pour ces différentes raisons, la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable a émis un avis favorable sur l'adoption de ces crédits, mais elle restera néanmoins vigilante. Mes chers Mes chers collègues, je vous rappelle que le temps de parole attribué à chaque groupe pour chaque discussion comprend le temps d'intervention générale et celui de l'explication de vote. Par ailleurs, le Gouvernement dispose au total de vingt minutes pour intervenir.

Monsieur le président, madame la ministre, madame la présidente de la commission de la culture, mesdames, messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, nous nous retrouvons ce soir pour examiner les crédits de la mission « Recherche et enseignement supérieur Domaine hautement stratégique pour la France, la recherche conditionne la compétitivité de nos entreprises et la performance de notre économie. Je le dis régulièrement, elle constitue également un formidable levier de développement économique et social pour nos territoires. L'enseignement supérieur est quant à lui cette porte ouverte sur le monde pour nos jeunes, ce guide chargé de les accompagner vers la réussite. Plus largement, il constitue le socle de la diffusion du savoir et, bien sûr,, de la recherche. On peut donc se satisfaire que la mission interministérielle « Recherche et enseignement supérieur » soit l'une des mieux préservées de ce budget 2019. Par-delà la ventilation et l'ampleur des lignes budgétaires, on retiendra que l'augmentation de ce budget est de 549 millions d'euros, pour un total de plus de 25 milliards d'euros.

je veux saluer les efforts accomplis par tous les acteurs dans la mise en place de la plateforme Parcoursup, qui, pour sa première année, a donné satisfaction. Raccourcissement du calendrier, mobilité intra-académique, ou encore présentation de l'offre de formation : plusieurs pistes d'amélioration ont déjà été envisagées.

enregistre une hausse non négligeable de 166 millions d'euros. Il marque ainsi la montée en puissance du plan Étudiants, dont l'objectif majeur est cher à notre commission de la culture puisqu'il s'agit de réduire l'échec en licence. L'effort budgétaire s'accompagnera d'une amélioration incontestable des conditions de vie étudiante que nous devons souligner. Pour la première fois, le coût de la rentrée universitaire a été significativement réduit d'une part, avec la suppression de la cotisation de 217 euros au régime de la sécurité sociale des étudiants ; d'autre part, avec le paiement à date des bourses. Pour la première fois aussi, la contribution vie étudiante et de campus, la CVEC, a été collectée. Si notre commission a émis des réserves sur les 95 millions d'euros budgétés, je crois que nous pouvons vous faire confiance, madame la ministre, pour que l'argent de la vie étudiante reste bien à la vie étudiante dans la loi de finances rectificative pour 2019. Il faut le reconnaître : ces changements sont loin d'être négligeables dans la vie et le budget d'un étudiant. L'année 2019 engage par ailleurs nos universités dans une double dynamique qui doit être poursuivie : d'une part, l'affirmation de l'autonomie des établissements, à garantir l'adaptation de l'offre de formation aux conditions locales ; d'autre part, l'incitation au regroupement, au sein des pôles de compétitivité, des contrats de site ou des projets de recherche collaborative. C'est une démarche indispensable face aux nécessités du temps. Je souscris pleinement à cette ambition qui consiste à développer le rayonnement international de nos universités, notamment au niveau européen. Le processus de Bologne a posé les bases de l'espace européen de l'enseignement supérieur, a harmonisé les systèmes nationaux et généralisé une division en trois cycles impliquant une reconnaissance réciproque des qualifications. Le système européen des crédits favorise la dimension internationale des formations supérieures, et c'est bien. Pour autant, l'université de demain doit également mieux s'inscrire dans son environnement régional. dans son environnement régional. Je pense notamment à nos universités d'outre-mer, qui ont vocation à davantage coopérer et échanger avec les pays de leur bassin géographique, au niveau aussi bien de la recherche que de l'enseignement supérieur. J'en viens maintenant à la recherche, qui se voit, elle aussi, portée avec ambition par ce budget. En effet, les montants alloués aux programmes de recherche du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation progressent nettement par rapport à la loi de finances pour 2018, pour atteindre 8,66 milliards d'euros en autorisations d'engagement et 8,76 milliards d'euros en crédits de paiement. Je voudrais particulièrement souligner l'inscription des 205 millions d'euros destinés à sécuriser le développement du lanceur Ariane 6. Le Centre spatial guyanais, qui a opéré en septembre dernier le centième tir d'une fusée Ariane 5, devra, avec ce nouveau lanceur, relever le défi d'une concurrence internationale accrue. Mon collègue Laurent Lafon, que je salue, que j'ai accompagné en Guyane en avril dernier, sera certainement d'accord avec moi visiter le Centre spatial guyanais vous donne un sentiment étrange, celui que, dans un autre temps, tout n'était qu'une question de volonté. C'est un sentiment assez surréaliste, entre la technologie la plus pointue et les disparités qui existent sur le reste du territoire. Alors, je dois le dire : lorsque les lobbies écologistes se précipitent en Guyane pour lutter contre tout projet industriel en expliquant que le territoire doit s'engager dans l'économie de la connaissance, je pense d'abord à nos 24 % de chômage et je souris avec amertume. selon une récente étude du cabinet Deloitte commandée par le WWF, la création d'un fonds de vitalisation de la biodiversité de 100 millions d'euros pourrait générer en Guyane plus de 10 000 emplois en quinze

il faudrait une volonté forte, comparable à celle qu'a déployée le général de Gaulle lorsqu'il s'est agi d'installer le Centre spatial guyanais en 1964. Très bien ! Mais en sommes-nous vraiment capables ? C'est là un chantier que je vous soumets, madame la ministre, et pour lequel vous m'aurez toujours à vos côtés : faire de la recherche française un moteur de l'économie de la connaissance en Guyane. De manière générale, il me semble essentiel d'articuler la recherche fondamentale et la recherche appliquée, et de favoriser l'interaction avec les entreprises dans les domaines d'avenir. La biodiversité, mais aussi l'économie bleue, l'économie circulaire ou encore le développement des biocarburants- en somme, tout ce qui converge vers la transition écologique -représentent une voie incontournable vers l'avenir autant que des filières d'emplois à structurer. notre groupe votera favorablement les crédits de cette mission. La parole Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, c'est avec une certaine gravité que je porte, au nom des chercheurs, de leurs syndicats et de plusieurs sociétés savantes, devant vous, une grande inquiétude devant le décrochage de la science française. D'année en année, la part du produit intérieur brut que la France consacre à la recherche ne cesse de diminuer. Elle était de 2,23 % en 2015 et elle devrait être de 2,19 Non seulement l'objectif ambitieux d'une part de 3 % du PIB s'éloigne inexorablement, mais son écart avec les taux de nos voisins ne cesse de s'accroître. Pour ne prendre que deux exemples, les dépenses de recherche de la Belgique rapportées à son PIB ont dépassé celles de la France en 2012 et ne cessent de progresser ; celles de l'Allemagne se trouvent quasiment au niveau de 3 % du PIB. Plus grave encore, les dépenses de recherche et développement des industries de la construction spatiale et aéronautique sont en forte baisse, de 3,2 %. Ce désengagement a des conséquences directes sur l'emploi des chercheurs dans ces domaines, en baisse de 1 %. À terme, c'est toute la capacité de recherche et d'innovation de notre pays qui est menacée. Au XVI siècle, Jean Bodin affirmait : « Il n'y a richesse, ni force que d'hommes. » La maxime s'applique avec encore plus d'évidence au domaine de la science : il n'y a pas de recherche sans chercheuses et sans chercheurs. Or les opérateurs publics voient leurs effectifs se réduire inéluctablement. Certes, dans les documents budgétaires produits par le Gouvernement, les plafonds d'emplois semblent préservés, mais, pratiquement, ils ne sont jamais atteints et il devient impérieux de nous interroger sur leur sincérité. Je salue la qualité de l'analyse budgétaire produite par notre collègue Jean-François Rapin, rapporteur spécial de la commission que le coût des mesures salariales décidées par le Gouvernement n'est jamais intégralement compensé et que les opérateurs de la recherche sont donc obligés de réduire leur masse salariale pour équilibrer leur budget. Ainsi, pour le CNRS, le coût supplémentaire du financement du seul glissement vieillissement-technicité, le fameux GVT, est évalué, pour le budget de 2019, à 25,3 millions d'euros. Il impose au CNRS de réduire son recrutement de cinquante chercheurs et de le porter à un niveau historiquement bas, qui compromet la crédibilité des concours et, en amont, la pérennité de nombreuses filières de l'enseignement supérieur. En deux ans, les effectifs du CNRS ont diminué de 375 équivalents temps plein. La baisse est de plus de 1 000 postes depuis 2011. Je partage totalement ce que fait observer Jean-François Rapin dans son rapport spécial : « Alors que notre pays cherche à attirer des chercheurs, la baisse des effectifs envoie un signal singulièrement négatif. » J'ajoute que la fuite vers l'étranger est devenue la seule issue possible pour une génération de chercheuses et de chercheurs qui se sent sacrifiée. Cette saignée a des répercussions sur la capacité de la science française à maintenir son rang. Ainsi, les financements obtenus par les équipes françaises pour le programme-cadre pour la recherche et l'innovation de l'Union européenne étaient encore de 13,5 % de son montant total, pour le cinquième programme, mais de seulement 11,3 % pour le septième, qui s'est achevé en 2013. De nombreux autres indicateurs attestent la baisse continue de l'influence de la science française. Je regrette vivement que vous donniez à votre ministère la seule ambition de l'accompagner. À cet affaiblissement de la capacité d'action des opérateurs publics s'ajoutent des choix stratégiques discutables, qui concentrent davantage les aides apportées à la recherche privée sur un dispositif, le crédit d'impôt recherche, ou CIR, qui mobilise plus de 6 milliards d'euros, pour des résultats que, désormais, la représentation nationale considère comme difficilement quantifiables. Je note que le nouveau fonds pour l'innovation et l'industrie, destiné à « garantir la souveraineté scientifique et technologique de notre pays et de son développement économique », répond à un totalement différent de celui du CIR. Ses axes stratégiques sont définis par un conseil de l'innovation, ses programmes confiés à des responsables chargés de leur mise en oeuvre, chaque action faisant l'objet d'une convention et d'un rendu évalué. C'est le fonctionnement normal adopté par tous les pays pour orienter et maîtriser leurs aides à la recherche privée. Il faut se demander pourquoi il ne s'appliquerait pas au CIR. Comme la recherche publique, l'enseignement supérieur souffre d'un désinvestissement de l'État dont les conséquences catastrophiques se mesurent notamment sur le taux d'encadrement des étudiants, qui ne cesse de diminuer. Comme pour les opérateurs de la recherche, les universités sont dans l'impossibilité d'atteindre leurs plafonds d'emplois. Ainsi, pour la période 2013-2016, seuls 76 % des emplois notifiés aux établissements ont effectivement été ouverts au recrutement. Dans un contexte de forte poussée de la démographie estudiantine, cette contraction ne permet pas d'améliorer l'accompagnement pédagogique, qui était pourtant l'un des objectifs de votre loi pour la réussite des étudiants. S'agissant de son application, il est très regrettable que votre ministère ne nous ait pas fourni un bilan complet de Parcoursup avant cette discussion budgétaire. Pourtant, les premières données très générales disponibles montrent que les bacheliers des filières techniques et professionnelles ont subi des discriminations sur lesquelles nous aurions souhaité vous entendre.

Monsieur le président, madame la ministre, mesdames, messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, « dans la lutte qui vient de finir,

Alors que l'intelligence artificielle est partout, de l'industrie à la santé, en passant par l'environnement, l'énergie et surtout la défense, il faut pouvoir placer rapidement la France en pointe des nations les plus influentes en ce domaine. Madame la ministre, vous avez dévoilé le 28 novembre à Toulouse la « stratégie nationale de recherche en intelligence artificielle », qui fait sienne cette ambition. Ce plan va bénéficier, au cours des quatre prochaines années, d'une enveloppe de 665 millions d'euros de la part de l'État, montant qui grimpera à un peu plus de 1 milliard d'euros pour la période 2019-2022. Si le signal est fort, ce secteur continuera néanmoins à voir ses cerveaux fuir à l'étranger, où les chercheurs français sont parfois les plus courtisés. Pour inverser cette tendance, il serait urgent de revaloriser les carrières des enseignants-chercheurs, notamment dans l'intelligence artificielle. Dans son rapport, Cédric Villani propose d'ailleurs de doubler le montant de leur salaire, et ce dès le début de leur carrière. Malheureusement, vous semblez exclure définitivement cette modalité et je serai vigilante à ce que d'autres voies soient trouvées pour lancer ce chantier de la revalorisation salariale. de la culture a estimé que le doublement du montant des primes de trois chercheurs sur quatre s'élèverait à 20 millions d'euros pour le CNRS et entre 30 millions et 35 millions d'euros pour l'ensemble des établissements publics à caractère scientifique et technologique. telle réforme ambitieuse serait de nature à renforcer la compétitivité de la France. Autre point de vigilance que je veux soulever : le manque de transparence sur le soutien de l'État aux domaines de recherche jugés prioritaires. La concomitance de nombreux dispositifs et d'annonces parallèles fait qu'il est quasiment impossible d'évaluer le soutien financier réel de l'État aux recherches considérées comme prioritaires, et ce d'autant plus que la plupart de ces financements ne sont pas liés à la mission « Recherche et enseignement supérieur Globalement, l'augmentation de crédits demandés au titre des programmes « Recherche » de la présente mission est de 2,4 % en autorisations d'engagement et de 2,9 % en crédits de paiement, ce qui traduit une ambition pour la recherche française qui reste en deçà de nos espérances. Alors que l'on connaît l'importance stratégique de la recherche et développement dans la croissance économique, le groupe du RDSE regrette qu'un effort supplémentaire n'ait pas été fait afin d'approcher l'objectif Europe 2020, qui a pour ambition de porter, à cet horizon, la part de la recherche et développement à 3 % du PIB. Or, d'après les indicateurs, en 2019, cette part sera seulement maintenue au niveau de 2018, soit 2,5 % du PIB. Je regrette également que l'évolution des crédits à la hausse sur le volet « recherche » soit uniquement captée par les programmes du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, alors que les programmes dépendant d'autres ministères verront leurs moyens au mieux stagner, au pire diminuer. Nous nous interrogeons sur la soutenabilité d'une telle politique à moyen terme et sur son implication sur les programmes en question, comme ceux qui visent à promouvoir la recherche culturelle et la culture scientifique et technique, avec, en son coeur, Universcience, dont le budget diminue une nouvelle fois. Même au sein de la MIRES, dont le budget se voit consolidé, nous ne pouvons ignorer l'impasse budgétaire dans laquelle se trouvent certains organismes de recherche, qui ne bénéficient pas des financements adéquats pour mener à bien les plans qui leur sont commandés- CEA, INSERM ou IFREMER. Parallèlement, la réforme de l'ISF a fait chuter les dons « d'au moins 50 % », selon France générosités, notamment en faveur d'organismes de recherche qui peuvent être fortement dépendants de ces contributions, comme le CNRS. le mécénat, la Cour des comptes ne traite malheureusement pas du mécénat des particuliers, mais je rejoins la rapporteure pour avis pour dire qu'il est nécessaire de trouver une solution pour le favoriser, afin de retrouver le niveau des montants dont bénéficiaient les opérateurs de recherche les années précédentes. du plan Étudiants, 123 millions d'euros supplémentaires doivent y être consacrés afin de répondre aux nouveaux défis de notre système, notamment l'afflux d'étudiants. Toutefois, ces nouveaux moyens risquent surtout d'être absorbés par la progression naturelle de la masse salariale et des dépenses. de la culture, une fois que les établissements se seront réellement acquittés de leurs charges incontournables, ne resteraient plus que 26 millions d'euros pour lancer des actions véritablement nouvelles en 2019. C'est trop peu Je rejoins le rapporteur spécial pour dire qu'il faut renforcer le pilotage des dotations des universités, généraliser le dialogue stratégique entre le ministère et les autorités académiques pour aller vers un pilotage plus fin des ressources des opérateurs. Mes chers collègues, même si ce projet de budget comporte des points d'inquiétude- que j'ai évidemment cités -relatifs à l'investissement de la France dans la connaissance et la recherche,

Ce budget, en troisième position dans le budget général de l'État, connaît une hausse de plus de 5 % en deux ans, et atteint désormais un montant de 28,17 milliards d'euros en crédits de paiement dans le projet Avec une part de 2,27 % du PIB, nous nous rapprochons de l'objectif européen de 3 %, mais nous sommes encore loin derrière les puissances technologiques que sont la Corée du Sud, Israël et le Japon. La mission est composée de sept programmes, dont le programme 142, « Enseignement supérieur et recherche agricoles ». Nous mesurons son importance

Formations supérieures et recherche universitaire », « Recherche spatiale ». S'agissant de ce dernier programme, madame la ministre, une grande partie de l'augmentation des crédits est fléchée vers le remboursement des dettes de la France envers envers l'Agence spatiale européenne. Mais 205 millions d'euros sont budgétisés pour sécuriser le lancement d'Ariane 6 en 2020. La mission que nous examinons est stratégique. Le bon fonctionnement de notre écosystème d'enseignement et de recherche, conjugué au dynamisme de nos entreprises, est un élément indispensable pour permettre à la France de s'adapter et de prendre part aux changements qui déstabilisent les anciens modèles et anciennes rentes. Au sein de la nouvelle économie, qui est celle de la connaissance et de l'immatériel, la concurrence s'exerce désormais par l'intelligence, par la capacité à innover et à préparer l'avenir. La première des priorités, madame la ministre, reste l'augmentation du niveau de qualification. Si les conditions d'insertion des jeunes diplômés se sont dégradées compte tenu du resserrement du marché du travail, le diplôme reste le meilleur rempart contre le chômage. L'accès à la formation tout au long de la vie est la deuxième priorité de cette mission. Les connaissances acquises aujourd'hui ne nous seront plus d'aucune utilité dans cinquante ans. Que chacun soit en mesure d'exprimer le meilleur de lui-même, quels que soient son parcours et son âge : voilà notre ligne d'horizon

Nous partageons la volonté du Gouvernement de favoriser les passerelles entre les formations et les générations, de développer une culture du progrès, de l'émancipation et du rebond. Le numérique est une opportunité inestimable. La mobilité géographique reste une nécessité. Aussi, madame

du choix du Gouvernement de diminuer de 5 millions d'euros l'enveloppe consacrée à l'aide au mérite, pourtant fer de lance de l'émancipation pour bon nombre de jeunes talents issus de milieux défavorisés. C'est désolant ! La France, pays aux 68 prix Nobel, se classe au quatrième rang mondial dans le système européen des brevets, mais n'arrive qu'à la septième place dans la part mondiale de publications scientifiques, sous l'effet de l'entrée en scène de la Chine, de l'Inde et du Brésil. Le soutien du Gouvernement à la recherche est fondamental. Le crédit d'impôt pour la recherche représente les deux tiers du soutien public à la recherche et développement privés. Le plan, la création du fonds de l'innovation et le positionnement stratégique de la France en matière d'intelligence artificielle et de recherche spatiale viennent renforcer l'attractivité et le dynamisme de notre écosystème de recherche national. Au sein du programme 172, cinquante bourses « convention industrielle de formation par la recherche » supplémentaires seront financées en 2019, permettant de renforcer les liens entre recherche et entreprise. Le bilan de l'examen de cette mission est plus mitigé en ce qui concerne les dotations du programme 190, « Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables Les moyens ne semblent pas au rendez-vous, malgré votre volonté politique affichée de faire de la France un acteur stratégique de l'énergie hydrogène, ce qui n'est pas tout à fait dans l'air du temps.

d'accentuer l'effort de recrutement d'enseignants-chercheurs et de personnels pour les accueillir et les accompagner, et d'intensifier la reconnaissance de l'engagement pédagogique dans le supérieur Sur le premier point, il faut saluer l'ouverture, en deux temps, de 30 000 places en licence pour accompagner l'arrivée de nombreux jeunes dans le supérieur à la rentrée 2018. Si la massification de l'enseignement supérieur est une chance pour notre pays, elle soulève plusieurs défis, au premier rang desquels figure l'adaptation de notre système pour accueillir au mieux les étudiants. Si on prend comme postulat initial un investissement moyen autour de 10 000 euros par étudiant, il faudrait, pour 2019, une augmentation de 400 millions d'euros afin d'absorber parfaitement la croissance de la démographie estudiantine. Cette année, les établissements d'enseignement supérieur bénéficieront de 206 millions d'euros de crédits supplémentaires. Or cette hausse, amputée des dépenses contraintes- GVT et compensation de la CSG, notamment -et de la montée en charge de mesures déjà engagées en 2018, ne servira qu'à financer 26 millions d'euros d'actions réellement nouvelles,

Sans effectuer un bilan exhaustif de l'an I de Parcoursup, plusieurs constats peuvent néanmoins être dégagés : Parcoursup, en tant qu'outil d'affectation, a plutôt bien fonctionné, peu de jeunes se retrouvant sans aucune affectation à l'issue de la procédure mais Parcoursup, en tant qu'outil d'orientation, a-t-il bien fonctionné ? Bonne question ! Rien ne prouve que la capacité de la plateforme à affecter correctement les étudiants soit un gage d'une orientation réussie. Ce n'est pas parce qu'un candidat accepte,, une proposition de formation qu'il est satisfait de qu'un candidat accepte,, une proposition de formation qu'il est satisfait de l'intégrer, d'autant qu'il n'existe plus de hiérarchisation des voeux. C'est l'énorme différence entre une orientation choisie et une orientation subie. C'est pourquoi, madame la ministre, je vous demande de nouveau, à l'image de la plupart des syndicats étudiants, de conduire et de publier une enquête nationale qualitative, à partir d'un échantillon représentatif, pour connaître véritablement le degré de satisfaction des étudiants quant à leur orientation. C'est uniquement à cette aune que nous pourrons évaluer Parcoursup comme instrument au service de l'orientation. Dernier point de vigilance, le nombre élevé de candidats ayant quitté la plateforme interroge : même si une partie d'entre eux s'est indubitablement dirigée vers des formations non répertoriées sur Parcoursup, il est évident que d'autres ont tout simplement abandonné la poursuite de leurs études. Madame la ministre, avez-vous pu effectuer une analyse plus fine de ces candidats dits « inactifs » ? Il est impératif, vous le savez, de lutter contre cette forme de décrochage et d'être encore plus proactif afin de l'endiguer. En ce qui concerne le volet « vie étudiante », la poursuite des efforts engagés au cours du précédent quinquennat, notamment en matière de construction de logements- 60 000 d'ici à 2022 -, est une bonne chose. Il en est de même du gel du prix du ticket RU et celui de la suppression de la cotisation d'assurance maladie, qui accroissent le pouvoir d'achat des étudiants. d'achat des étudiants. Pour autant, le plafonnement du produit de la contribution vie étudiante et de campus, la fameuse CVEC, à 95 millions d'euros, alors qu'il en est attendu un résultat- estimé par vos services lors des auditions -d'environ 130 millions d'euros, pose problème. Bien que vous ayez annoncé que l'intégralité de cette contribution serait reversée à la vie étudiante, en l'état, tout dépassement du plafond abondera, on le sait, le budget général de l'État. Alors, pourquoi attendre ? Pourquoi ne pas prévoir d'ores et déjà un plafond suffisamment haut, de sorte que la totalité de la CVEC profite immédiatement aux étudiants ? En procédant ainsi, vous éviteriez de susciter une forme de suspicion autour de la finalité de la CVEC elle n'a pas vocation à alimenter, vous le savez, même temporairement et partiellement, le budget de l'État ! L'amendement porté par notre groupe a été déclaré irrecevable, mais vous, madame la ministre, vous pouvez augmenter dès maintenant ce plafond en toute transparence. Dernière inquiétude, loin d'être anodine : la hausse des frais de scolarité pour les étudiants extracommunautaires à la rentrée prochaine. Alors, allez-vous me dire, quel lien avec le PLF 2019 ? Outre que la méthode du Gouvernement pose question, notamment sur l'absence de concertation, cette annonce complètement inattendue suscite déjà un vif émoi et réveille des tensions au sein de la communauté étudiante, alors même que nous sommes en train de débattre du budget. Surtout, nous aimerions comprendre en quoi multiplier par plus de dix les frais de scolarité pour ces étudiants serait source d'attractivité comme vous le prétendez. Soyons sérieux, ce n'est pas la création de 15 000 bourses- et voilà le lien avec le projet de loi de finances pour 2019 : où sont les crédits ? -qui sera de nature à compenser l'effet d'éviction massif des étudiants extracommunautaires pour raison pécuniaire, qui constituent, de surcroît, la grande majorité des jeunes venant étudier dans le supérieur français. La Suède a tenté récemment l'expérience, le résultat a été probant : une chute drastique de 80 % du nombre d'étudiants étrangers fréquentant ses universités. Est-ce ainsi que vous voulez améliorer le rayonnement de la France ? Est-ce ainsi que vous voulez atteindre le chiffre de 500 000 étudiants étrangers d'ici à 2027 ? Si nous souhaitons collectivement renforcer l'attractivité de la France, cultivons son image, dynamisons son réseau culturel, continuons à développer des formations à la fois reconnues à l'étranger pour leur qualité et leur spécificité. Mais ne cherchez pas à décupler les ressources des établissements supérieurs aux dépens de certains étudiants étrangers, ou- pour paraphraser un article paru dernièrement dans un quotidien -à « attirer les plus riches et, en même temps, à écarter les plus pauvres Nous en reparlerons, madame la ministre, car, sur le fond et sur la forme, c'est incompréhensible et c'est inacceptable ! La recherche est fondamentale pour le progrès scientifique et le développement économique. Pour la deuxième année consécutive, nous nous félicitons de ce que le budget consacré

a comme premier pilier l'excellence scientifique, qui vise notamment à « soutenir les chercheurs les plus créatifs et les plus talentueux dans leurs travaux de recherche exploratoire ». Or, en France,

de son budget à hauteur de 2 millions d'euros. C'est pourquoi je soutiens l'amendement de ma collègue Angèle Préville, qui a pour objet de réaffecter les 2 millions d'euros à Universcience. Pour finir, j'aimerais aborder la recherche afférente aux énergies renouvelables. Dans une note sur les dépenses publiques de recherche et développement en énergie en 2016, le Commissariat général au développement durable a mis en exergue que, depuis environ une décennie, l'investissement public en la matière s'est érodé. En 2016, En 2016, il s'élevait à 913 millions d'euros, soit 5 % de la dépense publique en recherche et 0,05 % du PIB ! Quel constat effarant, dès lors que la transition écologique- surtout actuellement -est érigée en priorité cardinale.

de 433 millions d'euros pour le financement de la recherche sur l'énergie nucléaire, et seulement de 51 millions pour la recherche sur les énergies renouvelables, soit neuf fois moins.

Certes, la France occupe une place prépondérante dans certains domaines, comme la biomasse, mais il serait plus opportun que les crédits alloués à la recherche sur ces énergies soient augmentés drastiquement. De plus, un changement d'échelle est nécessaire, comme l'a préconisé la Cour des comptes. Madame la ministre, vous l'avez compris, nous relevons des points positifs,

est sérieusement remis en cause : dans cette période de fortes tensions sociales, la discussion générale sur le troisième poste budgétaire de la Nation est évidemment un moment particulier de l'examen de ce projet de loi de finances. Le budget 2019 a un mérite qu'il faut saluer : il tient compte de la très forte pression démographique sur le système universitaire français. Vous le savez, d'ici à 2025, la population étudiante aura augmenté de 21 % en l'espace de dix ans seulement. Pourtant, pendant des années, les moyens alloués à l'enseignement supérieur avaient été décorrélés du flux de nouveaux étudiants. Après une progression de 2,7 de 2,7 % l'an passé, l'évolution globale des crédits de paiement à hauteur de 166 millions d'euros cette année va donc dans le bon sens. La pérennisation des financements alloués au titre de l'indemnité compensatrice de la CSG constitue, à ce titre, une bonne nouvelle. L'augmentation des crédits ne règle pas tous les problèmes pour autant. Pour le groupe Union Centriste, la priorité des années à venir doit être la lutte contre l'échec universitaire. Parcoursup a le mérite d'apporter des premières réponses dans la lutte contre l'allongement du temps écoulé entre l'obtention du bac et celle de la licence. La France reste malheureusement l'un des rares pays de l'Union européenne où moins de 50 % des étudiants valident leur licence au bout de quatre ans, contre plus de 75 % en Allemagne ou aux Pays-Bas. Les dizaines de milliers d'années d'étude perdues chaque année par les jeunes dans le supérieur sont évidemment un gâchis humain, mais aussi un gâchis d'argent public. En raccourcissant la durée d'obtention des licences à trois ans et demi, notre pays pourrait accueillir les futures générations d'étudiants à moyens constants, sans dépenser un seul centime de plus. Les dispositifs d'accompagnement « oui, si » doivent ainsi être fortement encouragés, encouragés, notamment sur le plan budgétaire : nous y veillerons attentivement. Les expérimentations menées par certaines universités- je pense en particulier à Paris-Descartes -sur les années propédeutiques méritent également d'être soutenues. Ce raisonnement nous rappelle que la hausse des crédits de paiement n'est pas une fin en soin. La tentation d'évaluer le budget de l'enseignement supérieur par un prisme purement comptable nous a fait oublier qu'un budget en hausse n'est pas nécessairement un bon budget. Méfions-nous de l'« effet cliquet » qui nous pousse à saluer la croissance perpétuelle des nouvelles dépenses sans jamais nous interroger sur la nature des dépenses passées reconduites. La légitimité du financement, essentiellement public, de l'enseignement supérieur français est une exception occidentale qui dépendra directement des performances et des réponses que cet enseignement apporte à la société française. Un euro dépensé pour l'enseignement supérieur est-il un euro systématiquement utile ? Quelle insertion professionnelle garantit-il pour les jeunes ? Permet-il de répondre aux besoins de l'économie et aux qualifications d'avenir ? Voilà les vraies questions que le Gouvernement doit se poser. À ce titre, le Sénat interpelle l'État depuis plusieurs années sur la permanence de nombreux archaïsmes, comme la procédure de qualification du Conseil national Surtout, l'État ne peut plus éluder aucune réflexion majeure comme l'est celle de l'offre de formation. Notre groupe partage les interrogations du rapporteur pour avis de la commission de la culture sur la pérennité des filières dans lesquelles sont constatées des places vacantes. De plus, vous l'avez reconnu en commission, madame la ministre, la demande insuffisante des jeunes générations pour les filières scientifiques nous fait défaut : il y a une révolution culturelle à opérer et à construire avec le ministère de l'éducation nationale. Cette nécessité de réfléchir très attentivement aux filières que la puissance publique privilégie et soutient est rendue d'autant plus nécessaire que les besoins de l'enseignement supérieur seront exponentiels Le comité pour la stratégie nationale de l'enseignement supérieur a évalué le besoin de financement à 1 milliard d'euros supplémentaires chaque année d'ici à 2020 ! Ailleurs dans le monde, des moyens colossaux sont mobilisés. À quelques kilomètres de notre frontière, à l'École polytechnique fédérale de Lausanne, les post-doctorants bénéficient d'un crédit d'installation dépassant parfois le million d'euros. Ces chiffres donnent le vertige : alors que l'argent public se fait rare, que les prélèvements obligatoires sont déjà excessifs, que le Gouvernement actuel n'a aucune stratégie efficace pour réduire notre niveau de dépenses publiques, comment allons-nous financer un modèle universitaire français à la hauteur du rang que notre pays est en droit d'ambitionner ? Le Gouvernement a décidé de baisser de 8 % les droits de scolarité en licence cette année, après trois années de gel la ministre, laisser nos universités se développer sans ressources propres significatives ? Ces questions imposent des choix forts, bousculant les équilibres établis. De ce point de vue, nous ne sommes pas opposés, par principe, à une augmentation des tarifs des étudiants étrangers, à condition, bien entendu, qu'elle s'accompagne d'une politique ambitieuse pour l'octroi de bourses. En matière de recherche, nous nous réjouissons que ses crédits augmentent de 330 millions d'euros par rapport à 2018, et de près de 830 millions par rapport à 2017. Union Centriste, la revalorisation des chercheurs est une question essentielle. En plus d'assurer la formation de nos étudiants, les chercheurs sont ceux qui permettent, par les avancées scientifiques sur lesquelles ils travaillent, de trouver des solutions aux enjeux écologiques, économiques, sociaux, technologiques de demain. Il est donc essentiel pour notre pays que cette matière grise puisse exercer en France dans de bonnes conditions, et ce sur le long terme. Nous ne le répéterons jamais assez un pays attractif pour les chercheurs, notamment internationaux, est un gage d'attractivité global pour l'avenir. Le prix Nobel de médecine, François Jacob, soulignait très justement : « Longtemps, la puissance d'une nation s'est mesurée à celle de son armée. Aujourd'hui, elle s'évalue plutôt à son potentiel scientifique. » Garantir et développer le potentiel scientifique français, voilà le défi à relever pour les années à venir. Nous voterons donc les crédits de la mission « Recherche et enseignement supérieur », car le groupe Union Centriste considère que ce budget est une première étape pour y parvenir, à condition d'assumer les choix courageux qui nous font face désormais.

Pour ma part, je préfère commencer mon propos par des félicitations : félicitations à l'égard des chercheurs français, qui font partie des meilleurs du monde et sont reconnus au travers de nos 36 prix Nobel, dont notre lauréat en physique cette année, Gérard Mourou. Il y a juste une semaine, six ans après Curiosity, la sonde InSight s'est posée avec succès sur Mars : exploit de la NASA, mais aussi des organismes et chercheurs français, puisque l'instrument principal qui va étudier la structure interne de la planète, le sismographe SEIS, est français, et même val-de-marnais. C'est dire l'excellence de nos chercheurs, puisque la France consacre seulement 2,2 % du produit intérieur brut à la recherche et au développement, très en deçà de l'objectif de 3 % de la stratégie de Lisbonne. En période de coupes budgétaires, le groupe Les Républicains ne fera pas partie de ceux qui voient la coupe à moitié vide, et nous nous réjouissons que ce budget soit en hausse même si, pour être plus exacts, le chiffre annoncé devrait tenir compte de l'inflation. Mon propos se concentrera sur trois programmes principaux : le spatial, l'Agence nationale de la recherche, l'ANR, et l'énergie. Vous avez décidé, madame la ministre, de respecter les engagements budgétaires internationaux de la France à l'égard de l'Agence spatiale européenne, l'ESA. Il me paraît difficile de faire autrement. Notre accès à l'espace, les lanceurs, les satellites ne peuvent se concevoir et se développer que dans cette configuration. Je ne peux que vous demander une nouvelle fois, comme nous l'avions déjà fait avec Bruno Sido en 2012 dans notre rapport sur la politique spatiale européenne, que soit mise en place, dans les faits, une réelle préférence communautaire. L'Europe est la seule puissance spatiale au monde assez masochiste pour ne pas confier ses lanceurs et ses lancements aux entreprises qu'elle finance. Compte tenu de l'importance de la contribution de la France au budget de l'Agence je souhaite, madame la ministre, que vous arriviez à faire évoluer les choses. Je reviens sur l'une de mes anciennes préoccupations : les débris spatiaux. Depuis le premier Spoutnik, voilà plus de soixante ans, les missions spatiales se sont multipliées ainsi que les débris et les risques de collision avec des satellites devenus indispensables à la vie quotidienne de plus de 7 milliards d'êtres humains, même si ces derniers n'en sont pas toujours conscients.

Passons, maintenant, à l'ANR, qui avait été bien malmenée dans le précédent gouvernement et envers laquelle vous tenez des engagements pris l'an passé. La revalorisation de ses crédits de 34 millions d'euros devrait permettre de faire remonter le taux de sélection des projets présentés par les équipes de chercheurs. Avec 14 % de projets en 2017, on est encore très loin des 20 % de 2012. Certains de mes collègues, dont le rapporteur spécial Jean-François Rapin, demandent que sa dotation soit un peu plus importante pour permettre le financement de plus de projets. Pour ma part, je continue à recevoir des mails de chercheurs qui estiment que l'ANR constitue un échelon administratif inutile. En tous cas, il est certain que la procédure de sélection est lourde et complexe. J'ai lu, sur le site de l'ANR, que « des évolutions ont été apportées à l'appel à projets 2019 afin d'améliorer sa compréhension et optimiser les modalités de dépôts des dossiers et d'évaluation ». Comptez-vous, madame la ministre, évaluer ce nouveau processus ? Seconde question : savez-vous si des projets portant sur le chlordécone ont été sélectionnés l'an passé ? Les Antilles ne pourront sortir de cette pollution que si les recherches aboutissent, et je suis persuadée que vous en êtes convaincue.

Ce programme est décevant : il est en baisse de 7 millions d'euros en crédits de paiement, alors que l'on sait bien que les opérations de démantèlement et d'assainissement des installations nucléaires à l'arrêt sont prioritaires, d'autant plus prioritaires que, voilà quelques jours, le Président de la République vient de décider de l'arrêt de nouveaux réacteurs, alors qu'il s'agit d'une production décarbonée. La recherche française doit pouvoir avancer sur les nouvelles technologies, comme celle de l'hydrogène. Le groupe Les Républicains votera ce budget, d'autant qu'il se réjouit du fléchage des crédits sur la recherche contre les cancers pédiatriques, qui n'ont pas été évoqués jusqu'à présent.

Qu'on se le rappelle : baisse des crédits affectés à la recherche, mise en place d'une sélection par tirage au sort, création d'allocations sans contreparties, à l'image de l'aide à la recherche du premier emploi c'étaient de mauvaises mesures, qui ternissaient l'image et l'efficacité de nos politiques en matière de recherche et d'enseignement supérieur. Assurément, ces choix questionnables et polémiques sont derrière nous.

continuera en effet de connaître, lui, une évolution inférieure à celle du budget général de l'État, et surtout à celle des effectifs d'étudiants. L'ambition de montée en puissance de l'enseignement supérieur ne se retrouve donc pas suffisamment dans ce budget ; le plafonnement de la CVEC à 95 millions d'euros en est l'illustration.

colmater des brèches déjà béantes et renforcer certains axes, sans que se dégage une politique globale. Deux chantiers me semblent pourtant essentiels. Le premier est de savoir comment rendre la recherche plus attractive.

elle atteint péniblement 2 800 euros au bout de dix ans de carrière. Nous serons donc tous d'accord, je pense, pour dire que cela porte préjudice à l'attrait et au dynamisme de la recherche dans notre pays. Vous nous proposez, certes, d'inscrire 130 millions d'euros de crédits supplémentaires : ils permettront essentiellement d'améliorer le déroulement des carrières, de déployer le protocole PPCR, de financer le glissement vieillesse-technicité, mais ils ne s'attaqueront pas à la mise à plat du régime indemnitaire des enseignants-chercheurs. Le second chantier est, bien entendu, la lutte contre l'échec massif des étudiants dans les premières années de leur parcours universitaire. C'est le cancer de l'enseignement supérieur et de notre société ; il prouve que l'université peine à répondre à la massification continue et à préserver cette belle spécificité française du faible coût de l'enseignement supérieur. Notre collègue Stéphane Piednoir a rappelé que le taux de réussite en licence n'était que de 28 % et que le Gouvernement envisageait d'atteindre péniblement 30 % en 2020. Je me demande si ces maigres objectifs n'avouent pas un manque de volonté politique. Il en est de même avec le plan Étudiants : 206 millions d'euros ont été annoncés, mais moins de la moitié seront effectivement affectés au plan, puisqu'une partie servira à payer le GVT et à compenser la hausse de la CSG. Madame la ministre, votre budget devrait porter l'ambition de renvoyer aux limbes de l'histoire ces taux d'échecs massifs qui caractérisent de nombreuses filières de l'université française et de l'enseignement supérieur. Pour cela, il faut allouer des moyens importants à la réussite des étudiants, diversifier les modes de financement de l'université, affiner le dispositif Parcoursup, donner toute sa place aux établissements privés d'enseignement supérieur, mais surtout travailler- et je crois que c'est la clé -à l'articulation entre le lycée et la licence, entre le lycée et l'enseignement supérieur. Or, depuis deux ans, nous constatons au contraire que les deux ministères travaillent en parallèle plutôt qu'en partenariat. Ainsi, la loi ORE a été lancée avant la réforme du baccalauréat, dans un calendrier où l'aval se désintéresse de l'amont et où l'amont ne cherche pas à comprendre l'aval. Le défi est bien, et vous ne l'abordez pas de manière frontale : c'est celui du « bac-3/bac+3 Les Républicains, je voterai les crédits de cette mission, enrichis des amendements de nos commissions. Toutefois, je crois qu'il est urgent de se retrousser les manches et de s'attaquer aux problèmes structurels de l'échec et du décrochage qui marquent l'enseignement supérieur, et de travailler pleinement aux liens entre le lycée et la licence,

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, voilà plus d'un siècle déjà, le Premier ministre anglais Benjamin Disraeli affirmait : « De l'éducation de son peuple dépend le destin d'un pays. » Universitaire, j'ai pu, pendant toute ma vie professionnelle, constater combien notre jeunesse a du potentiel dès qu'on lui fait confiance, dès qu'on lui donne les moyens de ses ambitions. J'aime à imaginer que de grandes figures comme Curie, Lavoisier, Buffon, Pasteur, Pascal, Ampère, Poincaré et tant d'autres nous regardent ce soir, en espérant que la France puisse retrouver son rang de pionnier dans l'éducation et la recherche scientifique : par le truchement de coupes budgétaires, s'est inexorablement terni. Je tiens donc à saluer le fait que la mission « Recherche et enseignement supérieur » est la troisième mission du budget général de l'État, avec 28,1 milliards d'euros, somme en augmentation de 1,8 %. Pour ce qui concerne la recherche, le programme 193, « Recherche spatiale », voit son budget en hausse de 205 millions d'euros. Le programme 172, « Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires », est quant à lui rehaussé de 171 millions d'euros. Je salue l'effort fait par le Gouvernement.

que ce site représente 14 établissements, 63 000 étudiants, 9 000 chercheurs et enseignants-chercheurs, 135 000 publications par an et près de 15 % de la recherche en France. Sachant que la population du campus devrait passer de 31 000 à 46 000 jeunes d'ici à 2022, ce désenclavement devient urgent, pour les conditions de travail et d'études sur place, mais surtout pour le rayonnement de ce pôle d'excellence scientifique tricolore. Pour finir, je souligne que le déroulement de Parcoursup, s'il a été moins chaotique que prévu, reste à améliorer sur plusieurs points. Je pense à l'amélioration des informations données aux candidats, au raccourcissement du calendrier, ou encore à la mise en place d'un répondeur automatique pour les élèves et parents en quête d'informations.

C'est du bon sens que de mettre en avant la recherche et l'enseignement de notre pays. Mais le Gouvernement devra prendre en compte nos recommandations et nos réserves ; nous les avons formulées, non pas pour le plaisir de critiquer, mais bien pour garantir à notre pays un rayonnement éducatif et scientifique à la hauteur de son histoire et de ses ambitions.

Monsieur le président, monsieur le président de la commission des finances, madame la présidente de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication, messieurs les rapporteurs spéciaux, mesdames, messieurs les rapporteurs pour avis, mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, tenir notre rang dans la compétition internationale, jouer un rôle déterminant dans l'élucidation des grandes questions scientifiques, favoriser l'innovation, mieux former et mieux diplômer nos étudiants sont les piliers de mon engagement en tant que ministre. ou MIRES, pour 2019 sont la traduction budgétaire de cet engagement, défendu par l'ensemble du Gouvernement depuis plus de dix-huit mois. L'objectif, affiché dans la loi de programmation des finances publiques, d'une MIRES dépassant les 28 milliards d'euros à l'horizon 2020 est pour l'heure respecté. Le budget que j'ai l'honneur de vous présenter a vu ses crédits augmenter de 5,3 % en deux ans, soit 1,3 milliard d'euros supplémentaires, dans un contexte financier que chacun mesure dans cet hémicycle. L'année prochaine, le budget du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation atteindra près de 25,1 milliards d'euros, soit 549 millions d'euros d'augmentation. Sur le périmètre complet de la MIRES, la hausse sera de 500 millions d'euros, portant les crédits de l'ensemble de la mission à 27,9 milliards d'euros. Ces montants ne prennent en compte ni les crédits du programme d'investissements d'avenir, ou PIA, qui abondent les universités et les centres de recherche, ni l'effort consenti par les collectivités territoriales et les entreprises au financement de la recherche, de l'enseignement supérieur et de nos politiques en faveur de l'innovation. En matière d'enseignement supérieur, l'année 2019 sera prioritairement consacrée à la poursuite de la réforme du premier cycle, pour laquelle les équipes des lycées et des universités se sont formées, au service de l'orientation des jeunes, dans un continuum du bac-3 au bac+3 C'est un peu plus de 123 millions d'euros qui financeront, au travers du programme 150, des parcours personnalisés de réussite, ainsi que les mesures indemnitaires qui permettront de soutenir et de valoriser l'engagement des équipes, tant dans la mise en oeuvre de Parcoursup que dans l'innovation pédagogique.

Toujours afin de mieux accueillir nos étudiants, 55 millions d'euros seront dédiés non seulement à l'ouverture de places supplémentaires, mais aussi au développement de formations courtes à fort potentiel d'insertion professionnelle. 33 millions d'euros permettront de financer les places créées pour l'année en cours et 22 millions d'euros sont d'ores et déjà prévus pour ouvrir de nouvelles places à la rentrée prochaine.

sociaux et de santé, ou BIATSS, notamment ceux des services de scolarité qui se sont engagés pleinement dans la réforme. Cet engagement supplémentaire mérite d'être souligné devant le Parlement.

à la baisse ininterrompue des subventions versées à l'enseignement privé. Près de 2 millions d'euros ont été abondés en gestion l'année dernière et « soclés » dans le budget de cette année. Nous tâcherons de réaliser en gestion un nouvel effort de 2 millions d'euros. Parce que la réussite académique est indissociable des conditions de vie concrètes des étudiants, la question de l'accueil et du financement de la vie étudiante est au coeur des politiques qui seront conduites par mon ministère pendant l'année à venir.

fixé en loi de finances à 95 millions d'euros, a été établi sur le fondement des prévisions réalisées par les services du ministère. Comme nous nous y sommes engagés, ce plafond sera révisé fin de 2019, à l'occasion du projet de loi de finances rectificative : dès lors, le montant effectivement perçu par les écoles et les universités à la rentrée prochaine pourra leur être totalement affecté.

Le Gouvernement est parvenu, pour la première fois, à réduire de manière significative le coût de la rentrée universitaire, notamment par la suppression de la cotisation de 217 euros au régime de la sécurité sociale des étudiants et par la mise en place du paiement à date des bourses. En 2018, la rentrée universitaire a donc coûté 100 millions d'euros de moins qu'en 2017 à l'ensemble des étudiants et à leurs familles. En 2019, je veillerai aussi à ce que nous nous donnions les moyens d'aller plus loin dans l'autonomie des universités. Avant la fin de cette année, nous publierons l'ordonnance relative aux regroupements expérimentaux.

au développement de leur propre signature. C'est un élément fondamental de modernisation du pilotage des opérateurs du programme 150, et j'espère pouvoir le généraliser dès que possible. Comme vous, j'estime qu'il est nécessaire de soutenir les établissements dans leur stratégie,

aux yeux des étudiants internationaux. Au-delà du triplement des bourses, 10 millions d'euros ont été mis à disposition des établissements au titre du fonds « Bienvenue en France ». De surcroît, 10 millions d'euros du ministère des affaires étrangères

sont inscrits. De plus, les étudiants internationaux disposant d'un diplôme de master ou de doctorat pourront travailler en France sans être obligés de rentrer dans leur pays pour demander de nouveaux visas de travail. C'est donc bien une véritable politique d'attractivité pour les étudiants internationaux que nous souhaitons mener. effet, il est extrêmement important que nous prenions en considération les attentes de ces étudiants en matière d'accueil. C'est pourquoi nous allons travailler, notamment, avec Campus France pour définir ce label

Parce qu'elle est tout aussi prioritaire que l'enseignement supérieur, la politique de recherche et d'innovation conduite par ce gouvernement sous-tend également la construction de la MIRES 2019. Afin de faire face à une concurrence internationale renouvelée par le volontarisme, en la matière, de la Chine ou de l'Inde, mes priorités sont simples : soutien à la recherche fondamentale, mobilisation des forces scientifiques pour répondre aux grands défis sociétaux et renforcement du partenariat entre universités et organismes de recherche. Il me semble indispensable de renforcer les missions nationales des organismes de recherche en leur confiant des programmes prioritaires de recherche à l'échelle nationale, à l'instar du à l'instar du programme pour le climat ou du programme dédié à l'intelligence artificielle. Au total, 29 millions d'euros, issus de la MIRES et du PIA financeront le volet « recherche » de Ces financements monteront en puissance année après année pour atteindre, au total, 665 millions d'euros sur la durée du quinquennat. Ce travail devra être mené en encourageant l'excellence scientifique de demain. Ainsi, le CNRS recrutera 300 nouveaux doctorants d'ici à 2020 pour renforcer les laboratoires. Au service de cette ambition, le budget de la recherche augmentera de 2,5 % cette année, soit une hausse de près de 8 % en deux ans. Cet effort souligne le caractère stratégique de la recherche pour notre pays. Le programme 172 disposera d'une hausse de 171 millions d'euros pour s'établir à 6,9 milliards d'euros. En matière spatiale, le programme 193 sera établi à 1,8 milliard d'euros, en hausse de 205 millions d'euros. Nous travaillons activement à la définition de la préférence européenne pour les lanceurs, et le conseil informel de Madrid a permis des avancées en ce sens. L'observation des débris constitue également un enjeu de plus en plus important. Plusieurs leviers sont actionnés, avant, pour limiter par la réglementation la constitution de ces débris, pendant, pour surveiller l'espace et éviter les collisions, et après, pour se débarrasser de ces débris. Plusieurs projets sont en cours, notamment chez Thales Alenia Space, qui considère cette question comme un véritable sujet d'avenir. Parce que la santé est l'une des plus urgentes préoccupations de nos concitoyens, mon ministère consacrera 17 millions d'euros en gestion au financement des plans Santé, qui sont, pour la plupart, menés par l'Institut

collègues députés, à l'unanimité des suffrages, pour mobiliser et mieux coordonner la recherche fondamentale dans la lutte contre les formes les plus résistantes des cancers des enfants. Nous mobiliserons ainsi 5 millions d'euros supplémentaires par an pour mieux valoriser les travaux de nos chercheurs.

Au titre des méthodes, j'ai la conviction qu'il ne faut pas opposer le financement sur projet au financement dit « de base ». Il faut recourir aux deux procédés, et il faut les employer au bon niveau, quel que soit le vecteur.

correspond un engagement ferme de l'État en termes de crédits de paiement : 86 millions d'euros en 2019, soit 220 millions d'euros supplémentaires en deux ans.

Je renouvellerai aussi mon soutien aux initiatives vertueuses permettant d'associer le meilleur de l'initiative privée et le meilleur de la recherche publique. C'est pourquoi, en 2019, l'effort de 5 millions d'euros déjà réalisé en 2018 au profit des instituts Carnot sera reconduit. Après avoir régularisé la situation de la France auprès des organisations scientifiques internationales à hauteur de 300 millions d'euros en 2018, dont plus de 170 millions d'euros hors secteur spatial, mon ministère restera, en 2019, pleinement engagé dans le financement des très grandes infrastructures de recherche,

Nous devons projeter nos politiques et nos pratiques à l'échelle européenne, dans le cadre de la préparation du programme Horizon Europe, le premier programme mondial en matière de recherche.

La négociation nous a permis d'obtenir une orientation générale partielle conforme aux grandes lignes attendues. Je songe en particulier à la création de l'agence européenne de l'innovation de rupture, l'EIC, avec un outil spécifique permettant l'émergence de start-up et un outil d'accélération dont la majorité des moyens sera dédiée à la croissance rapide, en combinant plusieurs types de soutien financier.

Cet appel à propositions, doté de 30 millions d'euros pour six projets pilotes, permettra à des consortiums d'établissements français et européens d'au moins trois pays de bâtir les premiers projets pilotes des universités européennes. Dans ce cadre, la France apportera son soutien à hauteur de 100 millions d'euros sur dix ans à la constitution de ces projets. Bien sûr, j'appelle tous les établissements français qui le souhaitent à se saisir de cette chance sans précédent, pour voir les premières universités européennes émerger dès la rentrée 2019. Mesdames, messieurs les sénateurs, telles sont les principales priorités du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en perspective de l'année à venir et la façon dont elles sont traduites dans le budget de la mission « Recherche et enseignement supérieur

budget moyen. En effet, le taux de financement moyen des programmes, qui était de 487 000 euros

que l'urgence climatique est, bien entendu, une priorité absolue de ce gouvernement. C'est pourquoi nous avons d'ores et déjà ouvert un programme prioritaire de recherche.

qu'une agence de moyens fonctionne bien, il faut qu'elle ait un gros volume. Sinon, les taux d'insatisfaction sont trop élevés. Cela demande énormément de travail aux chercheurs,

par l'État, sera mis en oeuvre par voie d'appels à projets de l'ANR. Ainsi, tout doucement, le Gouvernement tend à considérer l'ANR comme une nouvelle agence de moyens pour financer des projets nouveaux, qu'elle confie à des opérateurs sans leur donner de moyens de

je soutiens la liberté de conscience et je n'ai rien contre l'enseignement privé, catholique ou quel qu'il soit. Toutefois, en tant que sénateur et membre de la représentation nationale, il est selon moi indispensable, quand on soutient des structures

En quelques années, depuis 2008, ce dernier a perdu 45 % de l'accompagnement accordé par l'État, alors même que les EESPIG ont passé contrat avec l'État pour atteindre un certain seuil de qualité.

le Gouvernement y est défavorable pour plusieurs motifs. D'abord, l'action n° 04 du programme 150 visé par cet amendement finance exclusivement les établissements d'enseignement supérieur privé à but non lucratif, c'est-à-dire les associations et fondations reconnues d'utilité publique et les syndicats professionnels. La participation de ces établissements au service public de l'enseignement supérieur est reconnue par la qualification d'établissements privés d'intérêt général. Un contrat est conclu par l'État avec chacun de ces établissements, pour définir les conditions dans lesquelles ils exercent les missions de service public de l'enseignement supérieur, dans le cadre d'une gestion désintéressée. Les établissements s'engagent notamment sur des actions à mettre en oeuvre en matière de politique sociale : exonération des droits d'inscription des boursiers de l'État et attribution de bourses complémentaires ou de prêts sur critères sociaux

en amont, afin que les jeunes puissent se déplacer et préparer leur déplacement pour rejoindre des formations qui ont encore de la place, mais ne sont pas situées sur leur lieu d'habitation.

Il y a là une vraie réussite, qui s'explique par plusieurs raisons. Tout d'abord, il s'agit d'universités à taille humaine, de petits modules, qui attachent un intérêt particulier au développement des étudiants,

Cela fait partie de la doctrine de l'Église. On peut donc y enseigner, comme à l'Institut catholique de Paris, le droit canonique ou, mieux encore, le code des canons des Églises orientales, matières estimables que j'aurais personnellement aimé étudier.

pour soutenir l'innovation dans ce secteur, en le dotant, modestement, de 20 millions d'euros.

À l'heure où le réchauffement climatique s'installe, où l'avenir de nos sociétés est à construire, où chacun sera amené à faire des choix de vie, de société, et des choix politiques, il est plus que jamais indispensable que tout un chacun soit en capacité de comprendre, de savoir, pour être un citoyen éclairé, averti et conscient des enjeux. C'est le gage d'une société apaisée. S'agissant de la transition énergétique, rien ne se fera sans l'adhésion pleine et entière de nos concitoyens

Nous nous devons de permettre à nos jeunes de découvrir qu'ils aiment les sciences, de cultiver le goût de la science, celui des expériences et de la recherche. Nous aurons besoin à l'avenir de techniciens, d'ingénieurs, de chercheurs. Il y aura donc des postes à pourvoir pour les jeunes ayant ayant reçu cette culture scientifique. Leurs études demanderont un investissement que sublimera la passion nécessaire à la réussite. Ainsi la culture scientifique est-elle indispensable à la dynamique économique de notre pays. Nous aurons besoin de solutions innovantes pour résoudre les problèmes actuels, qui s'apparentent à des défis. J'avais déjà déposé cet amendement l'année dernière. Vous aviez évoqué, madame la ministre, un groupe de travail. N'ayant pas été sollicitée, je

de réduire les crédits de la recherche duale, mais plutôt d'attirer votre attention sur l'importance de la recherche culturelle et de la culture scientifique. Quel est l'avis de la commission ? Ma chère

la CSTI ne se résume ni au seul budget de l'État ni au seul programme 186. Chacun des 16 organismes de recherche, sous la tutelle du ministère, y consacre 1 à 2 millions d'euros par an. Il en est de même qui concerne le programme 150, puisque 125 millions d'euros sont prévus au titre de la diffusion des savoirs et des musées. Le ministère finance directement chaque année la fête de la science à hauteur de 1,1 million d'euros. Vous le savez aussi, depuis la loi NOTRe, la CSTI non plus seulement une compétence de l'État, mais une responsabilité partagée avec les collectivités territoriales, notamment les régions. Universcience est évidemment une institution extrêmement importante au coeur de la CSTI,

Cet amendement, plus modeste dans sa logique de transfert que les deux précédents, vise à transférer 900 000 euros du programme « Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires » vers le programme « Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

donc peu accessible à la myriade de petites entreprises qui constituent aujourd'hui notre écosystème de jeunes studios travaillant sur des jeux plus modestes,

Les dernières informations communiquées par le ministère du travail, en octobre 2018, montrent que le nombre de demandeurs d'emploi en catégorie A de moins de 25 ans a diminué de 1 % en un an

qui concerne tous les jeunes âgés de 16 à 25 ans, dont le montant maximal est de 484,82 euros par mois,

et nos concitoyens sur la réalité des montants consacrés annuellement à cette recherche fondamentale. À la différence des pays anglo-saxons, qui présentent des financements au coût réel, intégrant la masse salariale des chercheurs travaillant à améliorer notre compréhension des mécanismes fondamentaux à l'origine des cancers les plus résistants chez l'enfant, la France n'affiche que des financements additionnels